Il y a eu ces dernières années et ces derniers mois beaucoup de débats, de propositions ou de projets de loi sur la ruralité, l'hyper-ruralité et l'aménagement du territoire. Nous avons assisté, bien trop souvent, à de longues déclarations de bonnes intentions, à des listes à la Prévert des besoins à satisfaire, déplorant la désertification de certains de nos territoires. territoires. Le constat est partagé : des pans entiers de nos territoires se sentent légitimement abandonnés par la République, puisqu'il est de plus en plus difficile d'assurer à leurs habitants les services essentiels auxquels chaque individu a droit. Alors que la vie à la campagne est de plus en plus attractive dans l'imaginaire collectif, y compris pour les jeunes, qui y voient la promesse d'une vie moins stressante et plus en phase avec leurs besoins physiologiques et biologiques, le manque de service public et d'infrastructures freine cet appétit de vivre autrement.

par ceux que l'on qualifie d'experts et par les pouvoirs publics, pour l'aménagement du territoire, qui soumettent les femmes et les hommes, les entreprises et les territoires aux règles du capitalisme mondialisé de mise en concurrence et de rentabilité. Or la ruralité ou plutôt les ruralités ne peuvent entrer dans ce moule libéral. Nous en tirons une conclusion simple : il faut reconstruire des politiques publiques respectueuses des valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité, des politiques fondées sur la notion d'utilité publique et d'intérêt général plutôt que sur celles de rentabilité et de rationalisation de l'action publique, de limitation des dépenses publiques et, donc, de mise en oeuvre de l'austérité budgétaire à tous les niveaux de nos collectivités. Oui, l'État a un rôle à jouer et une responsabilité spécifique, en tout point du territoire national. À travers ce prisme, le bilan de ce quinquennat est redoutable, parce que les logiques libérales mises en oeuvre par la droite au pouvoir-

c'est-à-dire regroupés afin d'être moins dispendieux pour les deniers publics. Je pense notamment à tous les regroupements hospitaliers, qui ont conduit à éloigner les patients des lieux de soins.

D'ailleurs, lors du congrès récent de l'Association des maires ruraux, en octobre dernier, dans mon département de la Loire, une motion a été adoptée à ce sujet, appelant à une application plus souple des règles nationales au regard de l'enjeu spécifique du maintien d'une école en zone rurale. L'État a organisé sa propre disparition à travers la perte d'ingénierie, qui est pourtant une ressource essentielle en zone rurale, en diminuant les moyens humains au sein des préfectures, notamment dans les dispositifs Obnubilé par la réduction des déficits publics, l'État a renoncé à sa présence sur l'ensemble du territoire national, créant ainsi des droits à géométrie variable. La construction des infrastructures a pris du retard. Des lignes de trains et des gares ont été fermées ; l'aménagement numérique s'est heurté au manque de rentabilité dans certains espaces. Le rapport annuel de la Cour des comptes a d'ailleurs corroboré les inquiétudes régulièrement exprimées dans cet hémicycle. Le plan France très haut débit est sous-estimé et, surtout, ne comporte aucun engagement contraignant pour les opérateurs, ce qui conduit à son inefficacité. C'est d'ailleurs le problème principal. Les politiques de mise en concurrence généralisées se sont doublées de politiques de privatisation des services publics dans différents domaines : La Poste, France Télécom, EDF, les autoroutes ... Alors que la France s'est construite sur un modèle d'aménagement en réseau et de monopole public, tout ce réseau a été démantelé au nom des dogmes européens de libre concurrence, au terme de politiques qui ont conduit clairement à la disparition des services publics en zones non rentables, et donc en zones rurales. C'est l'essence même de l'action publique qui s'est diluée au profit de la finance. L'État a renoncé à son rôle de stratège et à son rôle de garant de l'intérêt général, laissant infrastructures et services au libre arbitre des intérêts privés. Alors que notre pays peut s'enorgueillir de s'être construit par un maillage fin du territoire territoire par les services publics, tout cet édifice semble aujourd'hui fragilisé, ce qui met en cause l'égalité républicaine, en zone rurale comme en zone périurbaine. Cette remise en cause alimente directement le Front national, qui prospère sur le terreau des renoncements, des injustices et du sentiment d'abandon républicain, souvent bien légitime.

l'ensemble des territoires. Le principe même de péréquation en matière d'aménagement du territoire tend à s'effacer progressivement. Conjuguée à la refonte de la carte de l'intercommunalité dans les territoires ruraux, cette tendance a conduit à accentuer les inégalités territoriales entre l'urbain et le rural. Privés de services publics et de présence de l'État, les territoires ruraux souffrent peut-être plus encore de la baisse des dotations poursuivies par les différents gouvernements depuis des décennies. Là encore, l'iniquité est grande.

L'avenir des territoires ruraux pose pourtant des enjeux économiques, sociaux, mais également démocratiques. En effet, privés de moyens humains, financiers et techniques, les élus locaux ont de plus en plus de mal à assumer leur fonction, ce qui produit frustration et découragement. La construction d'intercommunalités géantes par le relèvement des seuils posé dans la loi NOTRe a profondément déstabilisé le monde rural. Le seuil de 15 000 habitants n'est pas adapté à de nombreuses réalités territoriales. Surtout, ces regroupements se sont opérés de manière autoritaire. n'ont pas été fondés sur le libre consentement et les projets partagés, mais imposés par les préfets au travers de la commission départementale de la coopération intercommunale, la fameuse CDCI. Ce mépris démocratique a engendré un sentiment d'impuissance. Des compétences de proximité ont été confiées à des échelons trop vastes et la démocratie y a perdu. Ces regroupements forcés ont également eu pour conséquence, faute de moyens et de savoir-faire, de confier de plus en plus de missions de service public à des entreprises privées. Si le président du Sénat, reprenant l'expression de l'Association des maires ruraux, souhaite « oser la ruralité », alors il faut aller au bout de cette réflexion et en tirer toutes les conséquences. Le temps n'est plus aux assises ou aux constats, nous avons de la matière, notamment l'excellent rapport produit sous l'égide de l'Assemblée des départements de France, l'ADF, par mon ami Jean-Paul Dufrègne, ancien président du conseil général de l'Allier. Ce rapport contient des propositions intéressantes et novatrices qu'il conviendrait d'étudier très sérieusement. Le temps maintenant doit être celui de l'action, pour ces territoires, mais surtout pour leurs habitants. Ces territoires sont riches de ressources humaines, d'innovation, de solidarité et d'aménités positives. Les politiques publiques doivent les soutenir, les accompagner, les développer. Il convient donc d'agir prioritairement dans quatre directions. Premièrement, il faut stopper ces regroupements intercommunaux contraints, et donc inefficaces pour les habitants comme pour les territoires. Deuxièmement, il faut en finir avec la politique de baisse des dotations alors que les collectivités portent sur leurs épaules l'essentiel des politiques d'investissement. Il y a urgence à sortir de ce cycle moribond des politiques d'austérité, qui conduisent au déclin économique et à la souffrance sociale, sociale, et à définir un plan pluriannuel d'investissements pour la ruralité. Troisièmement, il faut revoir nos principes d'aménagement du territoire pour garantir la maîtrise publique des réseaux de communication, qu'ils soient de transports ou numériques. La fibre, qui est l'infrastructure du XXI siècle, doit irriguer tous les territoires. Pour cela, il faut en finir avec les politiques de privatisations et être capables d'imposer l'intérêt général comme fil conducteur de l'action publique. déclarer un moratoire sur les fermetures de services publics en zones rurales, pour cesser de désarticuler l'armature de la présence publique, qui répond aux besoins des populations, mais surtout les sécurise dans leur vie au quotidien.

que tout ce qui se trouve en amont, comme le machinisme agricole, ou en aval, comme le commerce. Si les activités agricoles constituent un secteur structurant, nous devons envisager la ruralité dans son ensemble. Après des décennies d'exode rural massif qui ont entraîné un vieillissement de la population, nous vivons maintenant un exode urbain. Chaque année, 100 000 personnes quittent la ville pour la campagne ; elles étaient 70 000 à faire le chemin inverse voilà 40 ans. Nous sommes donc loin de la mort annoncée et de la désespérance chronique dans laquelle certains voudraient cantonner les zones rurales. Aujourd'hui, pour consolider les communes rurales,

d'une commune de 591 habitants a justement fait le choix de ne pas céder à la désespérance. En 1995, alors que l'unique classe de l'école publique était menacée par le faible nombre d'élèves, plutôt que de baisser les bras et voir les habitants quitter progressivement le village, le maire a ouvert un centre de loisirs municipal, au risque de passer pour un illuminé aux yeux des élus voisins et de ses concitoyens. Vingt ans plus tard, une habitante témoigne : « C'est formidable, cela faisait soixante ans qu'un bébé n'avait pas crié dans le hameau ». aujourd'hui, plus de 30 élèves sont scolarisés et le centre de loisirs accueille 280 enfants par an. De quelle commune s'agit- il ? Ce maire a touché le coeur du problème : la présence des services publics dans les zones rurales. Chacun peut clamer son attachement à la ruralité- voire à l'hyper-ruralité ...-, être en première ligne de la défense des communes rurales, elles ne vivront que par la relance des services publics. En effet, les urbains quittant la ville pour aller vers le milieu rural souhaitent- et c'est bien normal -y retrouver les services de la ville. Face aux fermetures d'écoles et à la disparition des commerces, des communes rurales de l'Oise ont fait un pari similaire à ce maire de Corrèze. Ils ont opté pour la création d'habitats publics, comme à Cramoisy, où le maire a permis la construction de dix-sept logements HLM. Mais dans un département où 52 % des communes ont moins de 500 habitants, 89 % des 692 communes ne sont équipées ni d'une halte-garderie ni, évidemment, d'une crèche. Comment attirer de nouveaux habitants sans offrir des commodités essentielles, par exemple en matière d'accueil de la petite enfance ? Passons des paroles aux actes ! Assez de doubles discours entre, d'un côté, les fermetures de gares, de liaisons SNCF, jugées trop peu rentables, de trésoreries ou de bureaux de poste et, de l'autre, la défense de la ruralité, des territoires, des communes. D'un côté, on démantèle les grandes entreprises publiques, qui organisaient la péréquation et faisaient en sorte que, même au fin fond de n'importe quel village, par exemple en Auvergne, ... Ah ! ... on avait accès au téléphone, à l'électricité. De l'autre, De l'autre, on veut nous faire signer des contrats de réciprocité pour organiser la « solidarité territoriale ». Autrement dit, on fait désormais peser sur les villes

La désespérance est réelle, il ne faut pas la nier, mais elle n'est pas inhérente à la ruralité, c'est une conséquence directe du libéralisme et des cures austéritaires imposées aux communes. On voudrait nous faire croire que les communes sont responsables de tous les maux, qu'elles coûtent et, surtout, qu'elles pèsent sur les finances de l'État. Pour certains aspirants à la fonction présidentielle- il y en a quelques-uns en ce moment ! -, les dotations aux collectivités ne sont qu'une ligne budgétaire que l'on peut sabrer pour réduire des dépenses publiques prétendument excessives. J'en profite pour rappeler que les collectivités représentent à peine 9 % du déficit public, mais, surtout, 70 % de l'investissement public. Or cet investissement est évidemment un levier pour la croissance et l'emploi. En moins de trois ans, les communes ont perdu plus de 10 milliards d'euros de dotations. Il y a urgence à desserrer l'étau de l'austérité qui les étouffe et, à plus forte mesure, dans les zones rurales. En octobre, l'Association des maires ruraux de France dénonçait un projet de loi de finances pour 2017 « ruralicide » et s'attaquait, à très juste titre, à un énième renoncement de ce quinquennat : l'abandon de la réforme de la dotation globale de fonctionnement,

Comme le rappelait Cécile Cukierman à l'instant, notre groupe avait déposé une proposition de loi visant à réformer la dotation globale de fonctionnement et ainsi réduire les écarts de DGF de base entre le rural et l'urbain.

Quatre années après, pas de réforme et un quinquennat qui s'achève sur une baisse continue des moyens des communes avec toutes leurs conséquences ! Au-delà des contraintes financières, l'existence même de communes en zones rurales est remise en cause. L'obsession des fusions et des regroupements irrigue les grandes réformes territoriales, NOTRe et MAPTAM pour n'en citer que deux. Pourtant, la commune, bien qu'étant de plus en plus menacée- certains voudraient même en supprimer 30 000 ! -, demeure le meilleur pilier de la ruralité, échelon privilégié de proximité démocratique. démocratique. Les communes rurales méritent autant d'attention que les communes urbaines ; aujourd'hui, elles reçoivent autant d'austérité ! Je rejoins les demandes de ma collègue Cécile Cukierman, il est impératif de stopper les regroupements intercommunaux, d'interrompre les baisses de DGF et de revoir les principes l'aménagement du territoire. Il faut un moratoire sur les fermetures de services publics en zone rurale, il est urgent et indispensable de mettre un terme au recul de l'État dans ces zones et de donner les moyens aux communes de mettre en oeuvre les services publics.

de la modification indispensable du système des ressources de nos collectivités, ce n'est pas ce que j'appelle avoir une vision d'ensemble. C'est raisonner à la petite semaine, en fonction de contraintes qui, malheureusement, n'avaient rien à voir avec un meilleur fonctionnement des collectivités.

La parole est à M. Michel Canevet, pour le groupe de l'UDI-UC.

La parole est à M. Joël Labbé, pour le groupe écologiste.

de taille, celui de la stabilisation des comptes de la Nation après la crise de 2008 et les plans de relance coûteux du mandat précédent. Notre déficit public avait atteint des sommets et nous devions retrouver une plus grande maîtrise de nos dépenses. Cela s'est fait de manière souvent trop brutale et le Sénat s'est régulièrement fait l'écho des inquiétudes des communes rurales et des départements à dominante rurale.

pour les espaces ruraux, de fournir à la population des services publics aussi essentiels que l'accès aux soins de proximité, au très haut débit ou à la téléphonie mobile

beaucoup de communes encore qualifiées de rurales se trouvent sur des territoires où elles bénéficient d'une dynamique métropolitaine. Ce phénomène croissant de métropolisation entraîne mécaniquement, sur les territoires concernés- communes rurales comprises -, le développement d'activités économiques génératrices d'emplois et de richesses. Mais il reste cette partie des territoires ruraux que notre collègue Alain Bertrand

et représente seulement 5,4 % de la population. Celle-ci est souvent touchée par le vieillissement, l'enclavement, la faiblesse des ressources financières et le manque d'équipements et de services. Ces territoires méritent une attention toute particulière.

et les zones de revitalisation rurale, malgré les problèmes de transition que pose l'actualisation de ce zonage. Les défis à relever pour nos territoires ruraux restent encore très nombreux. Nous espérons que les efforts engagés se poursuivront et s'accentueront. et s'accentueront. Mes derniers mots iront à l'agriculture, notre agriculture, qui est en grande souffrance. Un travail

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le groupe CRC nous invite à discuter, une nouvelle fois- me semble-t-il -, de l'avenir des communes rurales.

territoire, ne fait plus sens. Elle est aujourd'hui dépassée par le fonctionnement du " système territorial ", fait de centralités, de réseaux et de flux de personnes, de biens, d'activités ou d'informations, à toutes les échelles et en interaction permanente et évolutive. Désormais dépendants les uns des autres, les territoires recèlent des capacités et des besoins différenciés, qu'il est utile d'appréhender. Ce rapport portait sur l'hyper-ruralité et le problème dont nous débattons se pose plutôt, à mon sens, pour cette forme de ruralité que dans le cadre d'une ruralité appréhendée de manière globale, et qui serait caractérisée par une situation, des problématiques, des forces et des faiblesses communes. Au même titre qu'il n'est pas sérieux de vouloir aborder les problématiques des territoires urbains de manière globale, utiliser le concept de « zones rurales » comme prisme d'analyse, notamment en matière financière, n'a pas de sens.

d'après les premiers résultats présentés par Bercy, la situation financière des collectivités locales s'améliore par rapport à 2015, ... Non ! ... du fait de recettes de fonctionnement progressant deux fois plus vite que les dépenses correspondantes. Je cite le secrétaire En somme, tout irait bien ! Évidemment, les réalités locales sont beaucoup plus contrastées et hétérogènes. Au sein des territoires ruraux, comme urbains, coexistent des situations très différentes d'une collectivité à une autre, qui tiennent notamment à la richesse économique de chacune d'entre Des problématiques de charges de centralité et de portage d'équipements structurants peuvent se poser, de la même manière, à des communes rurales et à des communes urbaines. En cela, de gros bourgs ou des villes-centres peuvent cumuler un certain nombre de problématiques et difficultés communes, qu'ils soient situés en zone rurale ou en zone urbaine. Rappelons-le, selon l'INSEE, 95 % des Français vivent aujourd'hui dans des communes sous influence urbaine. Les Français ne sont donc plus que 5 % à habiter des communes en dehors de l'influence des villes. L'opposition entre urbain et rural continue pourtant d'imprégner les esprits, alors que les relations et les interdépendances, qui lient la plupart des villes aux campagnes l'augmentation des mobilités et des échanges pour le développement, l'accès au travail, à l'enseignement ou aux loisirs, sont de plus en plus fortes. C'est ainsi que les attentes de certains des habitants de ces nouvelles ruralités sont liées à leur origine urbaine. À ce titre, l'accroissement de la taille des intercommunalités, à la suite de la loi NOTRe, et le seuil minimal de 15 000 habitants engendrent des défis indiscutables et communs aux zones urbaines et aux zones rurales. parvenir, dans des intercommunalités regroupant parfois plusieurs dizaines de communes, à mutualiser l'ingénierie publique au service de politiques d'équipement ambitieuses. Il s'agit ensuite de faire face aux risques d'augmentation de la pression fiscale dans des intercommunalités regroupant parfois

Cette question de la fiscalité est justement un des éléments disqualifiant le cliché d'une seule et même ruralité. De nombreux rapports ont démontré la grande hétérogénéité des taux de fiscalité dans les territoires ruraux, en fonction du portage ou non par la ou les villes assumant des charges de centralité et de services publics locaux à destination de l'ensemble de l'intercommunalité, par exemple en matière scolaire. Lorsque ce n'est pas le cas, l'absence de charges de centralité importantes va bien souvent de pair avec une fiscalité basse, mais également avec de moindres besoins financiers de la commune. La question des différences de charges entre communes rurales, et donc des différences de besoins en matière de ressources, fut l'une des principales questions auxquelles les groupes parlementaires ayant travaillé à une réforme de la DGF en 2016 se sont attelés. Les conclusions de leurs travaux étaient sans appel

Il est certain que le mode de calcul de la dotation de base des communes, en fonction d'un coefficient logarithmique aboutissant à attribuer plus aux territoires les plus peuplés, présente des limites, sachant qu'il a été conçu sur la base de travaux d'analyse maintenant un peu anciens.

kilomètres de voirie, critère de superficie, etc. -ont pu être intégrées au fil des réformes de la DGF dans les modalités de calcul de celle-ci. En outre, certains territoires ruraux bénéficient de ressources relatives à des spécificités locales, locales, certaines impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, ou IFER, qui constituent parfois une part non négligeable de leurs recettes de fonctionnement. Enfin, et c'était bien l'objet de la réforme de la DGF

La baisse des dotations entamée en 2014 a demandé un effort important à l'ensemble des collectivités locales du pays, c'est indéniable. Les chiffres de l'exercice 2016 que j'évoquais en préambule montrent que les collectivités locales sont parvenues globalement

Par ailleurs, il convient de rappeler que les territoires ruraux bénéficient de deux dispositifs de soutien financier puissants qui n'ont cessé d'être renforcés depuis 2012. En premier lieu, la DSR, ou dotation de solidarité rurale, qui

1,35 milliard d'euros. Cette évolution a permis de prendre en compte l'extrême hétérogénéité des situations connues par les communes rurales, et d'atténuer largement l'incidence de la baisse des dotations pour les territoires les plus pauvres. Au total, 4 317 communes de métropole ont vu le montant de leur DGF par habitant augmenter entre 2012 et 2016. le FPIC, ou fonds national de péréquation des recettes intercommunales et communales, qui est passé de 150 millions d'euros en 2012 à 1 milliard d'euros à compter de 2016. Toutes les études le prouvent, ce fonds constitue un outil puissant au service de la diminution des inégalités territoriales, et a notamment joué un rôle significatif pour les territoires ruraux. L'autre contrainte financière à laquelle peuvent faire face certains territoires ruraux est celle de l'investissement local. Là encore, d'importants dispositifs ont été déployés afin de soutenir les communes rurales et d'éviter qu'elles ne soient fragilisées par les baisses de dotations.

destinés à l'amélioration du cadre de vie et à l'attractivité des territoires, à l'aménagement des centres-bourgs ou des secteurs plus urbains, ou bien à des opérations en faveur de la transition énergétique et de mise aux normes des bâtiments publics. L'effet de levier souhaité s'est révélé particulièrement efficace : 800 millions d'euros d'aides attribuées au titre du FSIL en 2016 ont engendré 2,4 milliards d'euros d'investissements supplémentaires, soit au total 3,2 milliards d'euros d'investissement public local. J'ajoute que 43 % des subventions ont été accordées à des communes de moins de 2 000 habitants, pour un cumul de 128 millions d'euros. Par ailleurs, toujours dans le cadre de ce fonds, 216 millions d'euros seront cette année fléchés

tous les leviers ont été activés par le Gouvernement pour soutenir et renforcer l'investissement local, et notamment celui des communes rurales. On est sauvé ! Tout va bien ! Au vu de ce tableau général, il est indéniable que le Gouvernement et le Parlement ont veillé à ce que le redressement des finances publiques n'ait pas pour conséquence d'affecter trop fortement les finances des communes rurales les plus fragilisées, tout en les amenant à s'intégrer dans des intercommunalités de nature à les aider à se consolider et à répondre aux nouvelles attentes de leurs habitants. La parole

les libertés et droits des communes, départements et régions. Ces transferts de compétences ont évolué en fonction des grands enjeux économiques et sociaux. Il s'agit réellement d'un partage des responsabilités entre l'État et l'ensemble des collectivités territoriales : comment gérer les services de proximité sur le terrain, maintenir les équipements publics, soutenir

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, avec la réforme territoriale, on a en réalité peu évoqué la commune et le rôle qu'on souhaite lui voir jouer dans le nouveau paysage institutionnel. Je veux à mon tour remercier nos collègues d'avoir demandé l'organisation dans notre assemblée de ce débat sur les communes en milieu rural.

celle qui se trouve très éloignée des grands centres urbains, avec de nombreuses communes rurales qui, dans de vastes territoires, assurent le maillage de la présence humaine. Il faut connaître ces communes pour bien comprendre les missions remplies au quotidien par des élus locaux quasi bénévoles : les services apportés aux habitants, la veille exercée sur la vie locale, l'entretien des villages, le cadre de vie, la réalisation de projets de proximité, la solidarité, le lien humain. Dans une société toujours plus complexe, ces communes apportent, à moindre coût et dans la proximité avec les habitants, des réponses qu'aucune autre collectivité ne peut apporter. Vouloir mesurer l'intérêt du maintien de l'échelon communal au seul critère de son nombre d'habitants Dogmatique ! ... qui méconnaît la réalité du terrain. Bravo ! Bien sûr, les choses ne sont pas figées et les communes nouvelles apportent, dans certains cas, des réponses efficaces à des situations locales. Il appartient aux élus d'en décider. Quant au couple commune-intercommunalité, il n'est pas redondant, il n'est pas concurrent, il est au contraire parfaitement cohérent et complémentaire. Alors, avec quels moyens

de 3 milliards d'euros de DGF sur les 33 milliards d'euros affectés aux collectivités locales. On voit bien qu'elles ne ruinent pas notre République Ces communes, madame la secrétaire d'État, ont pris leur part au redressement des finances publiques, ... Oui ! ... mais nous devons désormais leur laisser les moyens de faire vivre la ruralité. Nous devons donner aux bourgs-centres et aux petites villes-centres les moyens de conforter leur rôle de pôles de services et d'emplois et aux plus petites communes, les moyens de remplir leurs missions de service public de proximité.

En ouvrant le sujet de l'avenir des communes rurales, on pose en réalité la question de la ruralité de demain. Je veux le dire avec force notre pays a besoin de sa ruralité ; une ruralité habitée, vivante, accueillante ; une ruralité innovante et connectée ; une ruralité

madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la loi NOTRe a prévu des compétences obligatoires pour les communautés de communes, mais les concours de l'État vers les communautés de communes sont en baisse et, surtout, le mécanisme de péréquation horizontale, le FPIC, est particulièrement injuste. Ce mécanisme présente des inconvénients. Tout d'abord, il se trouve que des communautés de communes qui étaient bénéficiaires du FPIC sont devenues contributrices. Eh oui ! Plus grave encore, des communes faisant partie de ces communautés de communes- qui étaient par ailleurs, elles aussi, bénéficiaires et, pour certaines d'entre elles, assez pauvres et même très pauvres -doivent désormais reverser de l'argent ... Voilà ! Ce mécanisme est donc très certainement à revoir, afin de corriger les injustices qu'il provoque, notamment au niveau communal, lorsque des communautés de communes accueillent en leur sein une commune plus riche, sans que, pour autant, la richesse de la communauté de communes soit établie, et encore moins celle de chaque commune qui la compose. Ensuite, on peut être choqué par le déséquilibre des mécanismes des dotations

Permettez-moi une remarque : puisque le Conseil constitutionnel estime que les populations doivent être numériquement équilibrées lorsqu'il s'agit de définir les limites d'un canton, pourquoi ce principe ne s'appliquerait-il pas à

et les communautés de communes ou les communes percevaient et perçoivent le produit fiscal de l'implantation de ces établissements industriels. Désormais, il me semble que la voie de l'investissement participatif ouverte aux communautés de communes et aux communes serait de nature à fournir des ressources assez

patrimoniaux et se comporter un petit peu comme des entreprises. En résumé, on dégage les moyens que l'on peut obtenir avec les moyens dont on dispose ! Il nous semble important de dégager de nouveaux moyens dans une période difficile, où la disette de l'État est avérée depuis de nombreuses années, et nous avons besoin de continuer à investir

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, les petites communes rurales sont plus que jamais à la croisée des chemins. En tant que président de l'Union des communes rurales de la Loire, je vois tous les jours qu'elles sont victimes d'un effet de ciseaux dévastateur, très bien résumé par l'intitulé de ce débat qu'a souhaité le groupe CRC. Les moyens des communes rurales sont réduits à peau de chagrin ! Partout, nous voyons réellement l'effet de la baisse des dotations. Les maires, désormais, réduisent les services rendus aux habitants.

de loi de finances pour 2017 entérine, pour la quatrième année consécutive, la baisse des dotations de l'État aux collectivités territoriales.

François Hollande a décidé, cette année, de pondérer la pression supportée par les communes et les intercommunalités en la réduisant de moitié, il n'en reste pas moins que, en 2014, 2015 et 2016, l'effort financier consenti par le bloc communal a été considérable. Il faut bien sûr mettre cet effort en relation avec les nouvelles charges imposées par le Gouvernement aux collectivités locales, par exemple, avec la réforme des rythmes scolaires dont la part du coût restée à la charge du bloc communal est estimée à 70 %.

Leurs dépenses moyennes d'équipement par habitant, en 2013, s'élevaient à 406 euros, alors qu'elles n'atteignaient que 396 euros dans les communes de plus de 3 500 habitants.

Ce rapport démontre très clairement l'effet de redoublement qu'ont les différentes dotations forfaitaires sur les inégalités initiales de richesse fiscale, contribuant à figer les inégalités de dépenses par habitant qui en découlent. Les premières analyses sur la réforme territoriale soulignent déjà que les incitations budgétaires pour encourager le développement de l'intercommunalité ont favorisé l'engagement de dépenses nouvelles plutôt que la recherche d'économies d'échelle. Nous avons beaucoup parlé des moyens, mais les outils, eux aussi, sont de plus en plus faibles. Nos collectivités arrivent de moins en moins à assumer l'ensemble de leurs missions et sont de plus en plus souvent délaissées par les services déconcentrés de l'État. En outre, lorsque les maires participent aux conseils communautaires, ils réalisent qu'ils n'ont malheureusement plus grand-chose à arbitrer. Il n'est plus question pour les communes de décider ensemble, en fonction du contexte et des possibilités locales, des compétences qui seront mises dans le « pot commun c'est la loi qui fixe la liste, de plus en plus longue, des compétences communales qui doivent obligatoirement être transférées au niveau communautaire. Dans toute la France, nous voyons les communes se dessaisir de leurs compétences- si j'ose dire -au Alors que l'urbanisme était un domaine incontournable de la gestion des communes, le transfert aux communautés de la compétence relative aux plans locaux d'urbanisme illustre parfaitement cet effacement historique. Les communes rurales minoritairement représentées au sein du conseil communautaire n'auront plus aucun moyen

même si nous manquons encore de recul pour évaluer certaines réformes, j'ai bien peur que nous ne soyons en train de créer des usines à gaz qui découragent les maires ruraux et qui ne soient source d'aucune économie, bien au contraire ! La parole

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, depuis les années 2000, les territoires ont connu une série de réformes qui ont profondément chamboulé le paysage administratif et politique de la France, création de nouveaux cantons rarement en rapport avec les bassins de vie, la création de nouvelles régions, le transfert de compétences du département à la région, la création de nouvelles communautés de communes- le Sénat a permis de maintenir un seuil de 5 000 habitants en zone rurale -, la création des pôles

en milieu hyper-rural, a perdu près de 40 000 euros au titre de la DGF ; j'ai sollicité, depuis un an, une aide pour automatiser une station-service,

semblent constituer un nouvel outil intéressant. Ils seront financés par le FNADT, mais sans augmentation de l'enveloppe. Là est le problème ! L'étude réalisée par notre collègue Bernard Delcros montre que les contrats sont aussi financés par un tassement des fonds

faveur des territoires ruraux vont dans le bon sens, nous constatons une baisse des dotations, une diminution des crédits de paiement pour les fonds alloués à la ruralité, qu'il s'agisse du FISAC ou des ZRR. cas les réunions de ce comité interministériel à des effets d'annonce. Je suis donc très inquiet quant à l'avenir des territoires hyper-ruraux qui auraient besoin d'aides spécifiques, avec des crédits en augmentation, pour la réalisation de projets de développement afin d'éviter la désertification. C'est encore possible

des maisons de santé, développer le tourisme, notamment le tourisme social, avec des crédits de réalisation ou de réhabilitation, encourager l'implantation des entreprises avec la mise en place, par l'État, de ZRR et de zones franches pour une baisse des charges- c'est par le biais du guichet unique,

Sans moyens ni aides spécifiques, il en résultera une désertification. Il faut instaurer pour l'espace rural une véritable politique adaptée, prendre quelques mesures simples et les financer véritablement par des aides directes, telles que des subventions, et des aides indirectes, comme les allégements ou suppressions de charges, afin de rendre attractif le développement de l'économie

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens tout d'abord à remercier le groupe communiste républicain et citoyen d'avoir pris l'initiative de l'organisation de ce débat aujourd'hui. Il intervient en toute fin de session parlementaire, signe que, jusqu'au bout de la législature, la Chambre Haute aura pleinement joué son rôle constitutionnel de représentante des collectivités territoriales. Je veux d'emblée, dès l'introduction de mon propos, saluer l'engagement de votre assemblée autour des sujets qui intéressent les territoires. Je fais partie de cette génération d'élus locaux qui n'a connu qu'un État décentralisé, et qui pense que les solutions pour nos concitoyens s'élaborent aussi, et peut-être d'abord, à l'échelle locale. Puisque nous sommes appelés à nous revoir un peu moins souvent, permettez-moi de saluer l'implication du Sénat sur ces questions et la qualité de son travail législatif. De plus, au moment où s'ouvre le temps de la campagne présidentielle, je ne peux malheureusement que constater, j'imagine, comme vous, que les enjeux territoriaux peinent à émerger dans les débats nationaux. Or je suis convaincue que ces questions ne doivent pas rester le parent pauvre des prochaines échéances électorales, car lorsque l'on parle de collectivités territoriales, on parle en réalité du cadre d'organisation des services publics locaux et donc de la vie quotidienne de nos concitoyens. Il nous revient, chacun à notre place et avec nos convictions, de plaider pour que ces sujets émergent. Le débat qui nous réunit aujourd'hui permet de remettre en perspective l'ensemble de ces éléments et de redonner cette vision globale si chère au président Mézard. La réforme territoriale menée sous ce quinquennat, qui a permis de clarifier le « qui fait quoi

Les régions sont désormais d'une taille adaptée au concert européen et sont dotées de compétences stratégiques en matière d'aménagement du territoire et de développement économique. À quel prix ! Elles disposent d'outils puissants pour les assurer : le schéma régional de développement économique, d'internationalisation, dont l'entrée en vigueur est prévue en 2017, et le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Ils doivent constituer de véritables stratégies globales et cohérentes.

renforcés sur la question de l'ingénierie territoriale et sur le cadre de l'élaboration du schéma d'accessibilité des services publics. En outre, ils interviendront toujours dans les domaines de compétences partagées comme le sport, la culture ou le tourisme, pour lesquels ils conservent une échelle d'intervention pertinente.

la priorité était donc de leur donner des périmètres adaptés aux bassins de vie des habitants, qui sont les territoires de la vie quotidienne des Français.

rappelle que 85 % des périmètres soumis à la discussion ont été validés par les élus dans le cadre de ces commissions, qui ont donné lieu à une grande mobilisation des élus. Cela représente une réduction de 39 % du nombre des structures. Les intercommunalités pourront ainsi exercer au mieux les nouvelles compétences qui leur seront transférées : en 2017, la collecte et le traitement des déchets, même si, nous le savons, de nombreuses intercommunalités disposent déjà de cette compétence, l'économie et l'accueil des gens du voyage ; en 2018, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ; en 2020, de manière obligatoire, l'eau et l'assainissement- j'ai d'ailleurs bien entendu les préoccupations du Sénat à ce sujet. Ce renforcement des intercommunalités n'est pas un mouvement supracommunal. Je suis, comme vous le savez et comme vous me le reprochez parfois aussi, une fervente militante de l'intercommunalité.

En écho à ce que disait M. Delcros, je pense plus largement que la commune conserve toute sa place dans cette nouvelle organisation territoriale en tant qu'échelon de proximité et de solidarité. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité qu'elle conserve sa clause de compétence générale, contrairement aux autres niveaux de collectivité,

pays, même s'il ne faut pas sous-estimer les tendances lourdes qui la traversent, comme en témoigne d'ailleurs l'abstention grandissante, y compris lors des scrutins municipaux. J'ajoute, car je ne veux pas cacher ce point sous le tapis, tout en espérant un soutien actif d'un certain nombre de sénateurs et sénatrices, que la modernité d'un échelon a aussi à voir avec sa capacité à s'ouvrir aux femmes. Or je ne peux, comme vous tous, j'imagine,

Je sais que le renforcement de l'intercommunalité peut nourrir des craintes chez les élus municipaux. Au contraire, il me semble qu'elle permet une plus grande solidarité entre les territoires d'un bassin de vie, si variés soient-ils : territoires riches, pauvres, urbains, périurbains, ruraux. L'intercommunalité n'a pas vocation à opposer ces territoires. À cet égard, je suis une fervente partisane des pactes financiers et fiscaux qu'il faut élaborer et approfondir partout, car il n'est plus acceptable d'avoir des communes pauvres dans des intercommunalités riches. À mon sens, il s'agit d'un enjeu majeur pour les intercommunalités. Dans les différentes lois de finances, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs d'assouplissement, visant notamment les attributions de compensation, qui permettent d'établir des pactes financiers et fiscaux pour que la redistribution des richesses s'effectue aussi à l'intérieur des intercommunalités. C'est, je le répète, un enjeu important et une condition de leur réussite à venir, ainsi qu'une contrepartie du renforcement de leurs Cette ambition de solidarité, même si le Sénat en fait un constat contrasté, est également portée par les territoires métropolitains, qui n'ont pas qu'une vocation de moteur économique, mais qui doivent également relever le défi de l'inclusion avec les territoires auprès auprès desquels ils rayonnent spontanément. D'ailleurs, vous le savez, dans le cadre du pacte État-métropoles, le premier contrat de réciprocité ville-campagne a été signé entre la métropole de Brest et le Pays du Centre-Ouest-Bretagne. Les zones rurales ! M.

Certains estiment que le processus de fusion permet d'avoir des communes renforcées, plus efficientes, c'est-à-dire mieux à même de jouer le rôle essentiel d'échelon de proximité et de répondre à tous les besoins du quotidien des citoyens. Selon moi, ce dispositif a vocation à se développer. Il s'appuie sur des bases volontaires et la souveraineté de la décision continue d'appartenir aux conseils municipaux.

et, plus récemment, la loi Sido du 8 novembre 2016 ont permis de moderniser le dispositif des communes nouvelles pour le rendre plus attractif. Je vous rappelle qu'il s'agissait d'une initiative parlementaire transpartisane.

517 communes nouvelles ont vu le jour grâce à la fusion de plus de 1 700 communes historiques regroupant une population totale de 1,8 million d'habitants. Comme le relevait le rapport du Sénat sur le sujet, il s'agit là d'une véritable « révolution silencieuse ». au-delà des questions institutionnelles, cette réforme territoriale vise un objectif concret : maintenir partout et pour tous des services publics accessibles et de qualité et porter des politiques publiques qui encouragent le développement de nos territoires. Les communes, de par leur vocation de proximité, sont bien évidemment en première ligne pour relever ce défi.

grâce aux 1 500 contrats d'engagement de service public à destination des étudiants, au contrat de praticien territorial de médecine générale, à la modulation régionale du, mais surtout grâce à la création des maisons de santé pluriprofessionnelles.

Je sais combien les élus et les administrés sont attentifs à cette question, et je mesure tout ce qu'il reste à faire dans certains territoires. Sur ce sujet essentiel pour l'attractivité du monde rural- qui

je nous engage à continuer à explorer toutes les pistes d'amélioration, qu'elles concernent les dispositifs nationaux ou locaux. Je crois utile que ces dernières réflexions soient conduites à l'échelle des intercommunalités pour éviter les concurrences parfois très féroces que se livrent les communes pour attirer de nouveaux professionnels de santé. Nous ne réglerons pas cette question du jour au lendemain, et nous n'infléchirons pas des trajectoires démographiques lourdes en un claquement de doigts, mais la mobilisation des moyens et des énergies va dans le bon sens. Il faut poursuivre nos efforts.

Ils sont par ailleurs accompagnés dans leurs projets éducatifs de territoire, et les regroupements pédagogiques intercommunaux ont été favorisés, comme certains d'entre vous l'ont rappelé. Enfin les « conventions ruralité », apparues en 2014 et fortement amplifiées pour la rentrée 2016, donnent une meilleure visibilité pluriannuelle aux territoires ruraux en matière scolaire, dans un contexte de baisse des effectifs du premier degré dans certains territoires ruraux éloignés des pôles urbains, ceux dont vous avez évoqué la situation voilà quelques Je le rappelle, c'est aussi le résultat des efforts en matière de créations de postes dans l'éducation, conformément à l'engagement du Président de la République de créer 60 000 postes sur le quinquennat. J'entends aussi sur mon territoire qu'il faut maintenir les écoles rurales. Je souscris à cet objectif, encore faut-il qu'il s'accompagne d'une politique de recrutement dans l'éducation nationale qui soit aussi à la hauteur des besoins en zone rurale. Cet effort de proximité est également porté par les maisons de service public,

Comme vous le savez, il y a aussi, et j'y insiste, car c'est un sujet sur lequel les départements sont très actifs, les schémas départementaux d'amélioration de l'accessibilité des services au public, en cours d'élaboration conjointe par les départements et l'État. Leur objectif sera de préciser les « zones blanches » sur lesquelles des maisons de services au public seraient utiles, pour, à terme, couvrir ces zones afin de garantir, sur tout le territoire, un accès aisé à une maison de service au public. aux questions liées à la téléphonie et au numérique, qui sont également au coeur des discussions.

des coûts de construction des pylônes dans les 300 centres-bourgs encore en zone blanche. Par ailleurs, 1 400 communes seulement couvertes en 2G le seront en 3G d'ici à mi-2017, et ce par les quatre opérateurs. Enfin,

2022. Il s'agit d'un élément d'attractivité important pour les communes, notamment rurales. Le développement de ce plan se poursuit, et 50 % de la population sera couverte par une connexion très haut débit à la fin de cette année. faux ! Ces mesures constituent des engagements forts envers le bloc communal, notamment en milieu rural. Elles sont pour la plupart issues des travaux des comités interministériels aux ruralités, les fameux CIR, nombre de trois en 14 mois, et à l'origine de 104 mesures. Pour veiller à la bonne déclinaison locale de ces différentes mesures, le Gouvernement a mis en place les contrats de ruralité, dont j'ai cru comprendre qu'ils étaient salués à peu près unanimement sur les travées de cette assemblée. Ils mobiliseront les dispositifs de droit commun, mais bénéficieront également d'une enveloppe dédiée de 216 millions d'euros au sein du FSIL. Plus largement, la loi de finances pour 2017 témoigne de l'importance que nous accordons au bloc communal, et plus particulièrement rural. D'une certaine façon, les chiffres illustrent tout autant, et certainement plus concrètement que les principes, l'importance que nous accordons à nos communes rurales. Les collectivités ont pris toute leur part au redressement des comptes publics. Là, on est d'accord ! S'agissant

Oui, rapide ! ... autour duquel tournent un certain nombre de discours orientés. Il n'est pas vrai de dire que, dans le cadre d'un plan d'économies qui serait de 100 milliards d'euros à partir de 2017, les collectivités ne verraient pas leurs dotations baisser.

Puisque ceux qui revendiquent ces mesures drastiques d'économies expliquent dans le même temps ne pas vouloir toucher au financement de la sécurité du pays, pas plus qu'ils n'entendent remettre en cause les équilibres de la sécurité sociale, ce qui est une chimère, comment font-ils ?

Les dotations de péréquation au sein de la dotation globale de fonctionnement progresseront ainsi de 380 millions d'euros, soit un montant inédit : 180 millions d'euros pour la dotation de solidarité urbaine, la DSU, qui sera d'ailleurs rénovée et 180 millions d'euros- un certain nombre d'entre vous ont signalé l'importance de cet effort -pour la dotation de solidarité rurale, la DSR. Entre 2012 et 2017, la DSU et la DSR auront progressé respectivement de 53 % et de 60 %, ce qui représente 900 millions d'euros de renforcement de la péréquation verticale. C'est un effort considérable à destination des territoires les plus fragiles. Enfin, le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le fameux FPIC, sera maintenu à son niveau de 1 milliard d'euros en 2017, alors qu'il était de 150 millions d'euros en 2012. Nous avons repoussé sa progression

qui doit être affecté au FPIC, car, si la réforme territoriale a contribué, comme je le crois, à lisser un certain nombre d'inégalités entre les territoires par l'augmentation

pour dire qu'elle a aujourd'hui vocation à s'installer dans le temps dans les périmètres actuels, sauf à ce que les territoires, d'eux-mêmes, décident d'évoluer dans le cadre du droit commun. Au-delà de cette progression de la péréquation,

et les communes et intercommunalités. La seconde sera dédiée aux territoires ruraux et aux villes petites et moyennes, qui ont leurs propres difficultés et thématiques, et financera également la progression de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, dotation

somme. À question précise, réponse précise : sur 1,2 milliard d'euros, 216 millions d'euros sont consacrés aux contrats de ruralité ; 150 millions d'euros visent à alimenter le financement des actions dans le cadre des contrats État-métropoles ; 450 millions d'euros iront sur les grands projets que vous avez précédemment cités ; 384 millions d'euros viendront alimenter la DETR, pour qu'elle soit portée à 1 milliard d'euros. Compte tenu de la division par deux de la baisse des dotations et de la stabilisation des nouvelles intercommunalités à un moment où les élus entament leurs projets de mandature, ces très importantes mesures de soutien doivent permettre de dynamiser encore la reprise de l'investissement local, qui a été

Fort de ce constat, et en tenant compte du fait que nous disposons d'une enveloppe normée et donc fermée, un certain nombre de scenarii ont été proposés. Celui qui a été retenu dans le cadre de l'article 150 de la loi de finances pour 2016 était une proposition de réforme qui, en effet, visait à simplifier la DGF en la faisant reposer sur trois bases : une dotation forfaitaire, une dotation de centralité, une dotation de ruralité. Cette réforme était réputée

l'ambitieuse réforme territoriale menée par le Gouvernement depuis 2012 constitue une nouvelle étape dans le mouvement de décentralisation engagée depuis le début des années quatre-vingt. Notre organisation territoriale est désormais plus lisible, ce qui était l'objet de la clarification des compétences, ... Dites-le à Mme Lebranchu ! ... mais elle est également plus coopérative et plus solidaire. C'est ce qui caractérise, à mes yeux, l'« âge de la maturité » de la décentralisation. Dans cette volonté d'alliance, de coopération et de solidarité entre les territoires, les communes, et particulièrement les communes rurales, ont toute leur place, j'y insiste. Leur proximité avec les administrés fait leur force, mais elles sont également, et de plus en plus, placées dans une relation de complémentarité avec leurs intercommunalités, car c'est en partie à cette échelle, qui recouvre les bassins de vie de nos concitoyens, que peuvent se construire de réelles solidarités, qu'elles soient financières ou fiscales. Je veux vous le dire, je suis optimiste en ce qui concerne la relation entre les communes et les intercommunalités. Je la crois apaisée sur le terrain, et j'ai confiance en la volonté des élus de porter leurs projets communautaires, au service de nos territoires et de nos concitoyens, dans le respect des identités communales auxquelles nous sommes tous attachés. C'est un mariage

: 3. Débat sur le thème : « Quel rôle les professions paramédicales peuvent-elles jouer dans la lutte contre les déserts médicaux ? » ; 4. Proposition de loi visant à assurer la sincérité et la fiabilité des comptes des collectivités territoriales